La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 mars 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation ?… Le procès verbal est adopté. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner demain à seize heures trente une demande d’attribution de pouvoirs de commission d’enquête pour une mission d’information sur les modalités de constitution d’une société commerciale par la Ligue de football professionnel. Par lettre en date du lundi 25 mars dernier, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a fait savoir qu’elle souhaitait modifier l’intitulé de cette mission d’information, qui porterait désormais sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Il n’y a pas d’observations ? Il en est ainsi décidé. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels est parvenue à l’adoption d’un texte commun. L’ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur la proposition de loi rendant obligatoires les « tests PME » et créant un dispositif « Impact Entreprises rapport n° 420). Mes chers collègues, je vous rappelle que ce scrutin s’effectuera depuis les terminaux de vote.

Ce n’est ni une hypothèse ni un postulat ; c’est une affirmation, une injonction sans laquelle la justice ne peut tout simplement pas être rendue de manière équitable.

il s’agit d’admettre que l’un des fondements de notre État de droit est devenu en grande partie inopérant. Certains édifices s’effondrent non pas parce qu’ils sont mal conçus ou parce qu’ils subissent des pressions trop fortes, mais simplement parce que leurs fondations ne résistent pas aux constructions qui s’accumulent au dessus d’elles. Ce raisonnement vaut notamment pour l’économie. La complexité du droit applicable obère notre compétitivité. elle fait peser sur les dirigeants des incertitudes juridiques qui deviennent insupportables. Au risque financier s’ajoute le risque juridique permanent, et les dirigeants vivent dans le doute permanent d’être hors la loi. Le président de la délégation aux entreprises l’a parfaitement résumé dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi Nul chef d’entreprise n’est censé ignorer les 11 176 articles du code du travail, les 7 008 articles du code de commerce ou encore les 6 898 articles du code de l’environnement. » Tout est dit.

Le président Rietmann a su formuler une proposition d’action concrète pour répondre à ces angoisses qui minent notre économie. En demandant que chaque norme, réglementaire ou législative, nationale ou européenne, soit d’abord évaluée à l’aune de ses effets sur nos entreprises, et moyennes entreprises (PME), nous proposons une nouvelle manière de produire la norme. C’est bon pour notre économie ; c’est bon pour notre démocratie.

haut conseil agira davantage sur le flux de normes que sur leur stock. Cela n’est certes pas la panacée, mais cela représente bel et bien une avancée.

a défendus améliorent le texte de façon pragmatique, en respectant l’esprit du texte original. Le repositionnement du haut conseil à la simplification sous l’autorité du Premier ministre lui conférera un portage politique plus important. Cela lui permettra également de travailler de façon transversale,

chiffres du déficit public par l’Insee conforte ma proposition. J’aurais trouvé plus raisonnable qu’il en fût autrement. En tout état de cause, il serait bienvenu que le haut conseil à la simplification soit placé sous le signe de la frugalité. La réduction de la dépense publique est en effet indispensable pour préserver la compétitivité des entreprises. Pour alléger la pression fiscale sans alourdir notre dette publique, il faudra réduire les dépenses publiques, et pour ce faire, rien de mieux que ne pas en créer de nouvelles.

Je ne parle même pas de la perte de compétitivité à l’international, où nos grands groupes et nos PME doivent rivaliser avec des concurrents qui bénéficient d’une administration bien plus agile.

Que penser également des études d’impact qui accompagnent tout projet de loi depuis 2009 ? Rédigées par l’administration, à la fois juge et partie dans l’affaire,

Bien sûr, je mesure l’ironie qu’il y a à dénoncer l’inflation législative alors que nous, parlementaires, endossons une responsabilité évidente dans cette situation. Ainsi, en plus d’un indispensable changement de culture administrative, nous devons aussi nous atteler à construire une nouvelle façon de fabriquer la loi. Il est indispensable de pouvoir produire des normes nécessaires, simples et compréhensibles, qui auront été coconstruites avec les entreprises, et dont l’impact aura été mesuré bien plus finement qu’aujourd’hui. C’est l’objet du texte que nous nous apprêtons à voter, déposé par Olivier Rietmann et enrichi par notre rapporteure Elsa Schalck. Ainsi, les « tests PME », dont l’objectif est de mesurer concrètement l’impact des normes sur les PME, nous permettront de rattraper notre retard

Son statut de commission administrative comme son rattachement au Premier ministre lui garantiront un portage interministériel de haut niveau. Son rôle d’évaluation sera important. À cet égard, nous avons clarifié et sécurisé les procédures de consultation. Le haut conseil sera obligatoirement saisi en amont par le Gouvernement sur tout projet ayant une incidence sur les entreprises. entreprises. Il est évident que ce texte va dans le bon sens, en proposant des dispositifs pertinents. Il me semble toutefois également important de rappeler que, faute d’un véritable changement de paradigme à tous les échelons de la décision publique, nous risquons de nous retrouver dans quelques années

En attendant, et en espérant qu’il donnera l’impulsion nécessaire, le groupe centriste votera ce texte.

Ayant été moi même responsable d’une petite entreprise, je peux témoigner de cette lourdeur administrative. Ah ! Elle pose un problème d’équité entre les entreprises de différentes tailles : souvent, les petits patrons ne peuvent pas payer des experts juridiques, à la différence des grands groupes.

certes, les codes continuent à s’épaissir, mais c’est aussi parce qu’ils contiennent des règles qui ne sont plus en vigueur. Mentionnons également la tendance à ajouter dans les lois des recommandations non obligatoires. Ce phénomène, que les Anglo Saxons nomment, vient lui vient lui aussi gonfler nos textes. Ensuite, nous devons questionner les conditions dans lesquelles nous légiférons. Oui, l’inflation législative est réelle, et certaines lois sont mal faites, le Gouvernement en est le premier responsable : l’usage de la procédure accélérée, normalement permis à titre dérogatoire, est devenu systématique. Cette généralisation touche en particulier les projets de loi les plus importants, qui méritent pourtant un examen approfondi de la part des parlementaires.

il faut faire une nouvelle réforme pour corriger les défauts et oublis de la précédente. Et l’on viendrait ensuite s’étonner que les entreprises n’arrivent plus à suivre le rythme ? Par ailleurs, la simplification n’est trop souvent qu’un prétexte pour affaiblir les règles régulant l’insatiable appétit de profit du capitalisme. Ainsi, c’est en son

vous proposez de créer un haut conseil à la simplification pour les entreprises. Chargé d’analyser toutes les règles applicables aux entreprises tant en amont qu’en aval de la procédure législative, celui ci aurait un pouvoir politique considérable obligatoirement consulté par le Gouvernement pour tout texte législatif, réglementaire ou européen ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, il pourrait émettre un avis défavorable obligeant le Gouvernement à revoir sa copie.

conférer un tel pouvoir à ce haut conseil revient à lui offrir de fait une tutelle sur la fabrique de la loi. Or le pouvoir législatif appartient au Gouvernement et au Parlement, et seul le Conseil constitutionnel est compétent pour trancher les litiges Oui, il est important d’associer les entreprises lorsque nous travaillons sur des textes qui les concernent. Cependant, qui parmi nous ne le fait pas déjà ? Les entreprises ne disposent elles pas de puissants lobbys pour les représenter ? Pourquoi leur donner encore plus de pouvoir et leur permettre de bloquer les normes qui les gênent ? La création de ce haut conseil conduirait à une nouvelle réduction du pouvoir du politique sur l’économie. Or le rôle du politique est d’arbitrer entre des intérêts divergents ! En plus du développement économique, nous devons aussi tenir compte de l’intérêt des travailleurs ainsi que des conséquences des normes sur la nature, sur l’environnement ou sur notre culture. La composition de ce haut conseil pose aussi question : s’il est censé aider les PME et très petites entreprises (TPE), pourquoi avoir alors ajouté un siège pour les représentants des grandes entreprises ? (Medef) n’a t il pas déjà assez de pouvoir ? À l’inverse, pourquoi avoir refusé notre proposition d’ajouter des sièges pour les représentants du personnel, pourtant les plus à même de faire remonter les contraintes juridiques que vivent les salariés au quotidien ?

Soyons en fiers ! À l’inverse, ne faudrait il pas aussi se pencher sur la « sous transposition » de directives et de règlements européens par la France ? Ainsi, nous craignons que ce haut conseil ne soit un nouvel outil pour attaquer les droits des salariés et les protections environnementales. Je vous rappelle d’ailleurs, mes chers collègues, que ces dernières peuvent être de vrais atouts pour nos entreprises.

Oui, nous sommes prêts à travailler à des simplifications qui aideront nos entrepreneurs et notre administration, mais pas de cette façon. Dans de telles conditions, le groupe écologiste votera contre

Troisième proposition : faciliter les ruptures de contrat. Quatrième proposition : réduire les délais administratifs pour saisir les prud’hommes. Si c’est cela, le « trop de normes sociales et environnementales », ce sera sans nous, et nous combattrons de toutes nos forces la loi Pacte II

mardi dernier, nous avons achevé l’examen de cette proposition de loi, portée par notre collègue Olivier Rietmann, visant à prévoir les incidences de la norme sur les petites et moyennes entreprises. Ancien entrepreneur, je connais les difficultés propres à l’arrivée de nouvelles procédures administratives. J’entends bien la détresse de chefs d’entreprise confrontés à un changement de nature législative qui, soudainement, désorganise une structure avant tout humaine et peut compromettre momentanément les métiers de ces entreprises. C’est la raison pour laquelle j’ai cosigné ce texte dès son dépôt, parce qu’il répond, selon moi, à de vraies inquiétudes et parce qu’il permettra, à l’avenir, d’anticiper l’applicabilité de la législation. Il revient au législateur de s’interroger sur l’efficience de la loi sur le terrain. Nous ne l’avons que trop constaté, avec la réforme du zéro artificialisation nette (ZAN). L’inflation normative est souvent dénoncée sur nos travées. Si nous pouvons faire des efforts de simplification, nous n’échapperons pas à la création de nouvelles normes, compte tenu des enjeux environnementaux et des politiques d’adaptation aux changements climatiques que nous allons devoir mener, qu’on le veuille ou non.

Penser le risque juridique au plus tôt pour les acteurs économiques de notre pays me semble donc un très bon objectif, pour que la loi retombe, si j’ose dire, sur ses pieds. C’est ce que prévoit ce texte créant un haut conseil à la simplification pour les entreprises, suivant par là une recommandation de l’excellent rapport d’information

Je me félicite de l’augmentation des effectifs issus des PME, car ce sont elles qui rencontrent le plus de difficultés d’adaptation face à la norme. En outre, la simplification pourrait alléger un climat qui est assez morose dans nos PME et TPE, comme le montre une récente étude de la Améliorer la visibilité des normes, c’est apporter un niveau de confiance bienvenu, dans le contexte d’incertitude qui pèse sur l’investissement. Le haut conseil sera consulté en amont des différents projets de législation et rendra des avis comportant un « test PME ». Il aura aussi une mission d’évaluation des normes en aval, ce qui est fondamental ; j’y reviendrai. Grâce à l’article 1 , cette instance bénéficiera d’une dotation pour couvrir ses frais de fonctionnement et ses travaux. L’article 1 , introduit en commission, définit ses compétences.

Le « test PME » inclus dans ces avis sera défini comme « [l’]analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises », de quoi parfaire les études d’impact de nos projets de loi…

En aval, la revue régulière des normes législatives et réglementaires en vigueur sera remplacée par une mission d’évaluation précise des normes applicables aux entreprises, effectuée à la demande du Gouvernement, des commissions parlementaires ou sur la propre initiative du haut conseil. Cette démarche en amont et en aval est confortée par cette nouvelle version du texte. Elle présente l’avantage d’entériner un processus vertueux qui permettra non seulement d’évaluer les normes, mais également de les coconstruire, afin de viser un « mieux de normes Un ajout important en séance, au sujet de la surtransposition des normes européennes, suscite des interrogations. Il ne faudrait pas que cette rhétorique bien connue devienne un leitmotiv pour revoir à la baisse nos engagements environnementaux et sociaux. Certaines évolutions législatives ont leur vertu, ne le perdons pas de vue. Hormis cette dernière remarque, dans la perspective d’une plus grande efficience de la loi, je crois que nous pouvons nous rassembler pour voter ce texte utile. C’est une première pierre avant un projet de loi de simplification annoncé pour l’été. C’est donc avec une vraie

l’excès de normes, leur imprévisibilité, leur complexité pèsent négativement sur l’activité de nos entreprises. Le coût des normes est estimé à 70 milliards d’euros par an, soit 3 % du PIB. Les entreprises vivent cette inflation comme une somme toujours plus grande de contraintes qu’on leur impose, comme un véritable frein pour leur compétitivité. C’est pourquoi le Président de la République, lors de ses vœux pour l’année 2024, a annoncé vouloir simplifier les normes et réduire les délais et les procédures administratives. Les Français y sont largement favorables. Devant les entreprises de boulangerie, Bruno Le Maire a ainsi annoncé deux nouvelles mesures de simplification. Après la suppression des formulaires Cerfa à l’horizon de 2030, les entreprises n’auront plus besoin de déclarer les arrêts maladie à la sécurité sociale à partir de 2027. Le dossier d’arrêt de travail, fourni par le salarié et le médecin, suffira. À partir de 2027 toujours, les employeurs n’auront plus besoin de réimprimer l’attestation d’assurance chômage pour la remettre au salarié. Les informations transmises par le salarié à France Travail suffiront. Au total, ce sont des dizaines de millions de documents par an qui seront supprimés. Sobriété administrative se conjugue parfois au mieux avec sobriété environnementale. Madame la secrétaire d’État, vous avez de votre côté confirmé le lancement d’un « test CSRD » () pour les PME. Elles « pratiqueront » la norme pour faire part de leurs remarques auprès de l’Union européenne. Cela est fondamental. Après l’inversion de la courbe du chômage, après l’inversion de la courbe des émissions de CO2, soyons déterminés à inverser la courbe, ressentie comme exponentielle, de la complexité. C’est ce que vous avez proposé, monsieur Rietmann, avec Jean Pierre Moga et Gilbert Luc Devinaz, dans un travail remarqué, présenté en juin dernier. La proposition de loi que nous nous apprêtons à adopter en est l’une des traductions. Avant d’assister à la fin des débats sur le Ceta, les entrepreneurs finistériens qui ont participé jeudi dernier à la journée des entreprises organisée par le Sénat ont beaucoup apprécié les échanges. Nous le savons, les attentes sont fortes, alors qu’une grande loi de simplification arrive bientôt. Comme cela a déjà été dit, la France se classe au deuxième rang des pays où la bureaucratie est la plus complexe. Il existe un autre angle lié à la complexification administrative qui n’est pas suffisamment abordé : il s’agit de la souffrance au travail et du sentiment d’inutilité. Nous avons pu le constater avec mes collègues députés, avec lesquels nous menons un travail sur ces problématiques. De nombreux témoignages nous ont été adressés, tels des appels au secours : « Il faut arrêter de légiférer sans cesse

Mais simplifier, c’est compliqué. Les majorités qui nous ont précédés en savent quelque chose. Monsieur Rietmann, c’est la raison pour laquelle vous proposez de changer le cadre, le logiciel de l’administration. Le groupe RDPI soutient totalement cette ambition.

la réalisation de « tests PME » sur les textes ayant un impact sur les TPE et les PME, l’évaluation des normes par une autorité indépendante et le pilotage de la simplification confié à un haut commissaire. En séance, mardi dernier, nous nous sommes prononcés pour la création d’un haut conseil à la simplification pour les entreprises, qui sera non pas une autorité administrative indépendante, mais une commission administrative consultative rattachée au Premier ministre. Madame la rapporteure, nous saluons votre travail sur ce texte. Vous avez aussi voulu préciser que les membres de ce haut conseil désignés par le Premier ministre le soient sur proposition des organisations professionnelles représentatives, au niveau national et interprofessionnel. Nous y sommes favorables. Le haut conseil sera consulté sur trois types de textes : les projets de loi, les projets de texte réglementaire et les projets d’acte de l’Union européenne. Il a également été prévu que le haut conseil alerte en matière de surtransposition de normes européennes dans le droit français. Nous soutenons également cette proposition. Mes chers collègues, il nous faut, oui, simplifier, mais simplifier sans déréguler, simplifier sans complexifier davantage. Appliquons déjà les règles existantes, de façon homogène, en expliquant les règles que nous adoptons. Formons ceux à qui elles se destinent, avant de faire le procès de leur non ou mauvaise mise en œuvre. Il faut soigner la relation entre les administrations et les usagers, avec moins de documents et plus de proximité, moins de défiance et plus de confiance. Monsieur Rietmann, vous avez raison, il nous faut une nouvelle méthode, non pour nous mettre, nous législateurs, sous tutelle, mais pour mieux raisonner. Le groupe RDPI soutiendra donc logiquement ce texte important et attendu.

la présente proposition de loi vise à rendre obligatoires les « tests PME » et à simplifier le cadre normatif pour les entreprises, mesures portées depuis de nombreuses années, qui, prises isolément, semblent parées de beaucoup de vertus. Pour autant, leur définition, leurs objectifs opérationnels et leurs conditions de mise en œuvre ne semblent pas suffisamment précis pour répondre aux attentes non seulement des entrepreneurs, mais aussi de toutes les parties prenantes de notre tissu économique. Dans une vie antérieure, j’ai eu la chance d’accompagner des chefs d’entreprise et des dirigeants d’organisation professionnelle. Comme vous, je peux témoigner de leur engagement résolu en matière de responsabilité sociétale. Mes collègues Brigitte Devésa, Lauriane Josende

J’imagine que certains seraient tentés de répondre qu’il n’y en a que de mauvaises. Je crois que ce n’est pas la majorité au sein du Sénat. En tout cas, pour le groupe socialiste, les choses sont très claires : ce n’est pas le « moins de droit » qui nous préoccupe, c’est bien le « mieux de droit », avec l’objectif de simplifier sans déréguler, comme l’ont rappelé Christophe Chaillou et Gilbert Luc Devinaz lors de la discussion générale.

Dans le Morbihan, une a été mise en place, sur l’initiative des chambres consulaires, des organisations professionnelles et interprofessionnelles. Nous constatons que cette demande est véritablement portée par l’ensemble des acteurs économiques. Enfin, si le troisième principe de la transition énergétique est le soutien aux énergies

nous avons la possibilité de faire mieux correspondre les lois que nous votons aux réalités de terrain. L’avant dernier point, madame la secrétaire d’État, concerne le rôle des corps intermédiaires et le besoin de différenciation.

sa mise en œuvre opérationnelle, de la même façon que des interrogations subsistent sur les moyens qui seront donnés au haut conseil. Nous constatons qu’un engagement a été pris sur une dotation dédiée, mais au regard de l’enjeu et de l’ampleur des sujets, cela nous semble très nettement insuffisant. Cette proposition

pleine et entière, contribuant à l’accélération des transitions écologiques et sociales, qui sont des facteurs clés pour la compétitivité de nos entreprises, pour aujourd’hui comme pour demain. Les chefs d’entreprise, qu’ils soient chefs de TPE ou de PME, d’ETI ou de grand groupe, nous le rappellent chaque jour. Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendra. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le débat en séance la semaine dernière a mis en lumière une large convergence d’analyse entre les propositions de notre délégation aux entreprises et le Gouvernement. Cette concorde tient notamment au travail réalisé par la commission des lois, et en particulier par son président, François Noël Buffet, et par sa rapporteure, Elsa Schalck. Je souhaite tout particulièrement rendre hommage à son travail sérieux et efficace, qui nous a permis d’aboutir à ce consensus. Je tiens à remercier également le président du Sénat, Gérard Larcher, et Bruno Retailleau d’avoir permis l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de notre assemblée. Je remercie également l’ensemble des orateurs, de tous les groupes politiques, de leur soutien. Ce texte est le fruit d’un rapport d’information adopté à l’unanimité par la délégation sénatoriale aux entreprises et d’une initiative parlementaire transpartisane. Cette convergence est fondée sur un constat partagé : « Notre pays souffre d’une accumulation démesurée de normes ! » J’emprunte cette formule à la ministre Olivia Grégoire, dont je tiens à souligner la disponibilité et l’écoute. Loin de moi l’intention de vous froisser, madame la secrétaire d’État, mais je regrette sincèrement son absence aujourd’hui. Je souhaitais la remercier de vive voix pour le travail collaboratif, engagé ensemble, avec simplicité. Je forme le vœu qu’elle accompagne cette proposition de loi jusqu’à son adoption, le plus rapidement possible, à l’Assemblée nationale. Certains me diront que les dispositions de notre texte trouveront leur place dans les projets de loi dits « de simplification » annoncés récemment par le Gouvernement. Ce n’est pas la bonne voie, car nous n’avons plus de temps à perdre. C’est dès maintenant que nous devons couper le robinet des normes. Nos ETI, nos PME et TPE souffrent et nous demandent de passer à l’action très concrètement. C’est dès maintenant que nous devons produire des études d’impact solides et de qualité. Les exemples ne manquent pas d’études d’impact indigentes, voire muettes, dans les différents projets de loi. J’en prendrai un. L’article 23 de L’article 23 de la dernière loi Immigration confère aux entreprises la responsabilité de financer les cours de français, pendant les heures de travail, pour les salariés qui ne maîtrisent pas suffisamment notre langue. Une audition récente de la délégation sénatoriale aux entreprises nous informe que cela représente un coût compris entre 24 000 et 33 000 euros par salarié Cela ne figure pas dans l’étude d’impact de la loi, parce qu’aucun « test PME » n’a été réalisé. Comment appréhender un texte dans ces conditions ? La méthode n’est ni sérieuse ni respectueuse du travail parlementaire. C’est dès maintenant, enfin, qu’il faut rendre obligatoire le « test PME ». Il doit concerner toutes les entreprises, de la TPE à la grande entreprise. Madame la secrétaire d’État, c’est une urgence économique ! Le réarmement de nos entreprises en passe par là. Si nous voulons y parer et observer de rapides résultats, faites que l’examen de cette proposition de loi se poursuive à l’Assemblée nationale. Mes chers collègues, je vous invite à voter massivement pour ce texte, qui vise à conforter les entreprises dans la guerre économique,

Monsieur le président, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté vise à répondre à une préoccupation majeure pour nos chefs d’entreprise l’inflation législative qui, depuis des années, complexifie la décision, renchérit les coûts de fonctionnement et laisse le citoyen souvent abandonné dans le brouillard du droit. Nous partageons tous ici l’attachement à la compétitivité de nos entreprises, dans un monde où la concurrence est féroce et souvent déséquilibrée. Cependant, la proposition qui nous est soumise aujourd’hui, bien qu’elle vise à résoudre un mal français persistant depuis des décennies, ne semble pas être en mesure de régler ce phénomène. Dès 1991, le Conseil d’État formulait dans son rapport annuel sa profonde inquiétude devant une loi tendant à la logorrhée, de plus en plus incompréhensible pour nos compatriotes et, pour le dire franchement, pour le législateur lui même. Depuis 2002, le volume de mots du droit français en vigueur a augmenté de près de 100 %. Derrière ces chiffres, on trouve des entrepreneurs, des élus et des citoyens perdus dans la compréhension de leurs droits. Par ailleurs, ce gouvernement, dont on nous vantait l’expertise et le sérieux, a été celui de tous les records en matière d’inflation législative. Les conséquences de cette prolifération de lois et de règlements sont désastreuses pour nos entreprises. Le coût macroéconomique de la réglementation est estimé à des des dizaines de milliards d’euros chaque année, ce qui pèse lourdement sur la compétitivité et l’innovation. Notre classement au niveau mondial en matière de performance du secteur public est alarmant, témoignant du fardeau réglementaire qui freine notre potentiel économique. Les PME en particulier sont les premières victimes de cette norme excessive. Obligées de naviguer dans un océan bureaucratique, elles peinent à se développer et à créer des emplois. Malgré des initiatives gouvernementales et parlementaires, comme la mission dite « Balai » (Bureau l’inflation législative demeure et le Gouvernement comme le législateur peinent à mettre leurs actes en adéquation avec leurs promesses. De plus, l’éphémère conseil de la simplification pour les entreprises, version pilote du projet que nous avons à examiner, n’a vraisemblablement pas répondu au défi de la simplification du droit pour nos entreprises. La création d’un haut conseil à la simplification pour les entreprises ne nous semble, à première vue, ni nécessaire ni adéquate. On irait ainsi créer un énième comité Théodule, alors qu’existent déjà le Conseil national d’évaluation des normes et de nombreuses instructions réglementaires pour essayer de limiter cette graphomanie irrépressible du législateur. Nous pensons que c’est par une gouvernance raisonnée et coopérative du ministère de la justice, du ministère de l’économie et des acteurs économiques qu’une législation efficace peut émerger. S’il nous faut agir pour alléger le fardeau normatif qui pèse sur nos entreprises, cette proposition de loi n’est pas, à nos yeux, nécessaire. Ainsi, les sénateurs issus du Rassemblement national s’abstiendront. Madame

Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Je vous invite à insérer votre carte de vote dans le terminal et à l’y laisser jusqu’au vote. Si vous disposez d’une délégation de vote, le nom du sénateur pour lequel vous devez voter s’affiche automatiquement sur le terminal en dessous de votre nom. Vous pouvez alors voter pour vous et pour le délégant en sélectionnant le nom correspondant puis en choisissant une position de vote. Le scrutin est ouvert.

Voilà bien longtemps que le sujet de l’inflation normative était sur la table ; plus que jamais, il appelait de nos vœux, comme des vôtres, à une simplification. Nos voisins allemands, néerlandais, suisses ou britanniques avaient déjà mis en œuvre des systèmes ayant le même objectif de simplification

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd’hui le projet de loi constitutionnelle

au report des élections mais défavorables aux modalités de celui ci. Quel que soit le sentiment qui habite les Calédoniens, quelle que soit leur volonté – indépendance, abstention, attachement à la France

pour les élections locales. Je constate d’ailleurs que la liste électorale « référendaire » est plus large que la liste électorale « provinciale

Bien sûr, ces règles institutionnelles parfois paradoxales, en tout cas originales, ne s’opposent en rien au respect des identités des uns et des autres.

Aujourd’hui, nous participons tous à écrire une nouvelle page de l’histoire calédonienne. Cette page doit être celle de la stabilité : elle doit permettre aux Calédoniens et à tous les acteurs économiques et sociaux de ce magnifique territoire du Pacifique

Les accords précités ont introduit dans notre droit la notion de citoyenneté calédonienne, concrétisant le destin commun des communautés qui composent la Nouvelle Calédonie et vivent sur un même territoire.

L’histoire calédonienne nécessite que ceux qui sont de passage sur le territoire ne soient pas pleinement associés à son avenir. Cette affirmation est en soi discutable dans une démocratie dans laquelle on paie des impôts et dont on a la citoyenneté, mais,

du congrès de Nouvelle Calédonie. Celui ci est important en ce qu’il donne une majorité pour diriger la Nouvelle Calédonie. Par ailleurs, nous connaissons la symbolique du congrès,

Il s’agit donc de bien plus que de simplement voter pour des représentants locaux. L’enjeu électoral se conjugue, ici comme partout, à un enjeu de représentation, d’autant que le gouvernement collégial de la Nouvelle Calédonie est composé à la proportionnelle. depuis la révision constitutionnelle de 2007, seules les personnes inscrites sur les listes électorales au moment de l’accord de Nouméa de 1998 ont le droit de voter aux élections provinciales.

Nous ne proposons que le dégel du corps électoral, dans certaines conditions, pour les élections locales. Le corps électoral référendaire permet aux personnes qui ont vingt années de résidence en Nouvelle Calédonie de participer au référendum sans justifier d’une inscription sur les listes électorales à une période donnée.

Si le gel du corps électoral provincial n’excluait, lors de son vote en 2007, « que » 8 338 électeurs en 1999, soit 7,5 % de l’électorat,

Nous savons tous qu’en 2007, la volonté du président de la République et du gouvernement de l’époque était de mettre en place ce gel de façon transitoire. Mon prédécesseur Dominique de Villepin avait lui même précisé devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles ce gel ne valait que pour les élections provinciales de 2009 et de 2014. C’est bien sur le fondement de cette donnée que le Parlement avait alors voté pour le gel du corps électoral.

là d’une position politique que l’État assume pleinement pour tenir sa parole, engagée au Congrès que je citais, et non pas seulement d’une préoccupation d’ordre juridique. Il me semble important qu’au bout de trois ans de discussions

Je rappelle par ailleurs que le Conseil d’État a lui même considéré que l’importance actuelle de la restriction du corps électoral soulevait un doute très sérieux sur sa compatibilité avec les engagements internationaux de la France, alors que le processus défini par l’accord de Nouméa est achevé, les trois référendums ayant eu lieu. Le Gouvernement s’est donc engagé à corriger cette distorsion, qui n’est pas conforme à l’exercice du droit de suffrage sur un territoire de la République. La France est une démocratie. Le Président de la République et le Gouvernement ont toujours affirmé leur intention de procéder à un élargissement du corps électoral par une initiative unilatérale, celle du Parlement, si aucun accord n’était atteint avant la fin de l’année 2023. Je tiens à votre disposition les documents l’attestant, signés par les responsables politiques y compris indépendantistes. Cette initiative n’est donc en rien une surprise et l’on ne saurait jouer la montre contre le droit de suffrage. Il s’agit dès lors de définir un cadre stabilisé et équilibré. Là où les indépendantistes sont opposés au dégel du corps électoral, les non indépendantistes proposaient de retenir des durées de domiciliation comprises entre un et trois

On peut être contre cette proposition ; on peut aussi être contre le fait que des gens votent, refuser le suffrage du peuple pour choisir ses représentants locaux, mais alors ce n’est pas le projet d’un pays démocratique. J’ai plusieurs fois entendu les termes d’« accélération » et de « marche forcée

Il ne s’agit pas d’imposer un accord global sur la Nouvelle Calédonie. Le Gouvernement est attaché à l’autodétermination, dont il souhaite envisager les modalités avec toutes les parties, y compris les indépendantistes. Il est attaché à un accord global sur les institutions de la Nouvelle Calédonie, sur la définition de la citoyenneté, et il n’impose rien. trompons pas de débat : le Gouvernement veut juste que les Calédoniens puissent voter aux élections locales pour désigner les représentants locaux et participer, en Nouvelle Calédonie comme partout en France, aux élections.

paraître tautologique, mais ce n’est pas le cas en Nouvelle Calédonie. Prendre une décision, choisir tel ou tel candidat, se présenter devant les électeurs, savoir à qui l’on parle, pouvoir choisir son destin, être citoyen,

il s’agit de la répartition des sièges entre provinces au sein du congrès. J’entends ce que disent les élus non indépendantistes du territoire, leur démarche est logique.

D’innombrables réunions ont été organisées à Nouméa et à Paris. Plusieurs textes écrits, coécrits ou réécrits rendent possible un nouvel accord, fondé sur des modalités d’autodétermination, sur la citoyenneté calédonienne, sur les discussions économiques – elles sont dans tous les esprits – et, bien évidemment, sur le temps long, dans le respect des trois référendums.

Cela reviendrait à désavouer les votes précédents, et donc le suffrage, tout en créant une instabilité qui nuirait définitivement aux investissements et il y aurait en permanence une épée de Damoclès au dessus de la Nouvelle Calédonie. Écoutons les Calédoniens : l’incertitude actuelle bloque l’essor de leur territoire. Il faut que les investissements reprennent, que les services publics fonctionnent, que la santé soit garantie, que les cotisations et les impôts rentrent,

Jusqu’à présent, nous avons longuement discuté des perspectives de cet accord sans y parvenir. Près de trois années se sont écoulées depuis la dernière consultation. Le message que le Gouvernement adresse à la Nouvelle Calédonie est le suivant : avançons, ne bousculons pas les équilibres, proposons une solution de compromis sur la question du dégel du corps électoral sans préjuger d’un éventuel accord global. Le Gouvernement y est prêt et tend la main à tout moment. Il est de la responsabilité de l’État de garantir l’expression du droit de suffrage sur l’ensemble des territoires de la République. Nous le souhaitons toutes et tous, parce que nous sommes une grande démocratie. Les Calédoniens, souvent, nous démontrent que ce paradoxe existe dans ce magnifique archipel : parfois, plus on est

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’intérieur et des outre mer, cher Gérald, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis pour débattre au sujet d’un de nos territoires d’outre mer qui nous sont si chers. Le texte constitutionnel dont nous allons discuter concerne ce territoire, la Nouvelle Calédonie, dans lequel je me suis rendu avec mon collègue Gérald Darmanin voilà tout juste un mois, pour y dire l’engagement total de l’État et du ministère de la justice en particulier. J’ai pu en effet inaugurer le centre de détention de Koné.

La Nouvelle Calédonie est un territoire particulièrement attachant et j’ai pu constater la richesse des cultures qui y cohabitent. C’est aussi un territoire dans lequel le

Cette originalité était déjà présente dans la reconnaissance par l’accord de Nouméa d’une citoyenneté calédonienne. Il s’agissait là d’une innovation majeure, porteuse d’une forte charge symbolique. Cette citoyenneté se manifeste notamment par l’existence d’un corps électoral spécifique aux élections provinciales et aux élections du Congrès.

ou qui y résident depuis plusieurs décennies. C’est à ces Français là que je pense. Lors du déplacement en commun que nous avons effectué, nous avons rencontré beaucoup de Français, qui nous ont fait part de leur incompréhension et de leur frustration de ne pas pouvoir participer à la démocratie. C’est aussi bien sûr à nos règles que je pense, et particulièrement à l’article 1 de la Constitution, selon lequel la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, Je pense également à son article 3, qui pose clairement le caractère « universel, égal et secret » du suffrage, et qui affirme avec force que sont électeurs « dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Enfin, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame de façon solennelle : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. ce gel du corps électoral contrevient également aux obligations internationales de la France. L’article 3 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales affirme la nécessité d’organiser, « à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif

pouvait paraître « disproportionnée au but poursuivi », mais elle avait admis la conventionnalité du dispositif, qui s’inscrivait dans un processus transitoire et répondait à une situation très particulière. Cette décision aura vingt ans dans quelques mois. La situation démographique a largement évolué et la Cour pourrait être désormais saisie

Si les circonstances propres à la Nouvelle Calédonie sont toujours de nature à justifier l’existence d’un corps électoral spécifique, la compatibilité des règles en vigueur avec les engagements internationaux de la France est aujourd’hui plus qu’incertaine, alors que le processus défini par l’accord de Nouméa est désormais achevé. Les trois référendums d’autodétermination organisés en 2018, 2020 et 2021 ont en effet tous conclu au refus de l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle Calédonie. Aujourd’hui, plus de 40 000 de nos concitoyens peuvent voter aux élections nationales, mais sont privés du droit de vote aux élections du congrès et des assemblées de province. Parmi eux,

toutes ces personnes soient exclues de la démocratie calédonienne. Comme vous le savez, la priorité absolue du Gouvernement reste la conclusion avec les partenaires calédoniens d’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle Calédonie. C’est la raison pour laquelle, de manière inédite, il est prévu que l’entrée en vigueur du projet de loi constitutionnelle soit subordonnée à l’absence de conclusion d’un accord entre les partenaires politiques.

Il a, en outre, décidé de confier au Conseil constitutionnel le soin de constater l’existence d’un accord répondant à ces caractéristiques ; ce rôle s’inscrit parfaitement dans les missions déjà confiées Ce projet de loi constitutionnelle confie par ailleurs au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la révision constitutionnelle. En tant que garde des sceaux, j’ai conscience du caractère inhabituel de ce renvoi. Pour son application, la Constitution de la V République renvoie traditionnellement à la loi organique et à la loi ordinaire. Toutefois, vous l’avez compris : ce mécanisme n’est en rien une défiance, bien au contraire. L’intervention du pouvoir réglementaire est justifiée par l’urgence de la situation, le Gouvernement s’étant engagé à ce que les élections ne soient pas reportées au delà de 2024. L’esprit même de notre démocratie, chacun le comprend, ne permet pas de retarder ces élections, et impose un dispositif qui assure la plus grande célérité. Pour renforcer les garanties encadrant l’intervention du pouvoir réglementaire, le Gouvernement a fixé les matières dans lesquelles ce décret est susceptible d’intervenir la composition du corps électoral, les opérations de révision des listes et divers critères d’appréciation des conditions d’inscription. Il a également limité dans le temps cette habilitation : ce décret ne pourra être adopté qu’avant le 1 septembre 2024. qui concerne la possibilité de reporter la date des élections jusqu’au 30 novembre 2025 en cas de conclusion d’un accord entre les partenaires politiques, je serai plus bref. La jurisprudence constitutionnelle admet la possibilité de prolonger les mandats en cours des membres de l’organe délibérant d’une collectivité dans un but d’intérêt général. Toutefois, le législateur n’est pas libre : il doit évidemment respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle. Cela implique notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité jugée raisonnable. le report d’élections ne peut intervenir au delà d’un délai raisonnable de dix huit mois. En prévoyant un report au plus tard au 30 novembre 2025, le Gouvernement s’inscrit pleinement dans la ligne jurisprudentielle qui guide notre droit électoral. Mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du Gouvernement, j’ai l’honneur aujourd’hui de porter devant vous, avec mon collègue de l’intérieur et des outre mer dont je veux ici saluer le formidable engagement, ce projet de loi constitutionnelle. Je tiens à le rappeler avec force le destin commun de la Nouvelle Calédonie est dans les mains des Calédoniens eux mêmes. Si la priorité du Gouvernement demeure la conclusion d’un grand accord entre les partenaires politiques afin d’aboutir à une nouvelle organisation politique durable respectueuse des sensibilités de chacun et fidèle aux acquis de l’accord de Nouméa, il nous faut agir pour mettre fin à une injustice démocratique, qui prive de droit de vote aux élections au congrès et aux assemblées de province un électeur calédonien sur cinq.

je veux saluer tout particulièrement nos collègues de Nouvelle Calédonie, Georges Naturel et Robert Wienie Xowie, qui nous ont beaucoup aidés dans la préparation de ce débat, en s’attachant à nous donner une information précise sur la situation du territoire et en se faisant force de proposition. Monsieur le ministre de l’intérieur, vous l’avez dit : une page se tourne ; il faut en ouvrir une autre, comme en 1988 avec l’accord de Matignon, comme en 1998 avec l’accord de Nouméa. La stabilité et le devenir du territoire supposent que les représentants de toutes les

un souci d’équilibre, mais aussi que le Gouvernement joue un rôle actif dans les négociations.

à l’évidence, il ne s’agit pas de cela aujourd’hui. Si chacun admet qu’un cadre stable ne peut être posé pour la Nouvelle Calédonie que dans le cadre d’un accord, il n’est pas en notre pouvoir de donner le temps long que vous réclamez à juste titre, monsieur le ministre de l’intérieur, par un vote du Parlement.

Le texte qui nous est soumis ne porte pas une telle ambition. Il vise simplement à sortir du blocage du corps électoral qui fait que, en dehors des électeurs de statut coutumier, on ne peut plus accéder au vote aux élections provinciales. Il faut donc permettre le dégel du corps électoral pour en faire un corps électoral « glissant ». C’est bien la moindre des choses, car nous sommes arrivés à une situation qui écarte du vote non plus 7 % des électeurs, comme au moment de la révision constitutionnelle de 2007, mais,

– le garde des sceaux a rappelé qu’elle était fondée sur l’article 3 de la Constitution française – doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Elle ne l’est plus aujourd’hui, en raison de cette proportion très importante d’électeurs écartés des élections provinciales.

que la disposition de la Constitution qui gèle le corps électoral disparaisse. Je tiens à dire – il y a eu des incompréhensions à l’égard du travail de la commission des lois – que cette volonté s’est exprimée en commission dès la semaine dernière. Le choix d’un dégel permanent, irrévocable, irréversible, par abrogation d’une disposition constitutionnelle qui permettait le gel, est le choix de la commission des lois, comme il a été le choix du Gouvernement lorsqu’il

qui sont les plus importantes de Nouvelle Calédonie. Par conséquent, le Gouvernement nous propose d’intégrer à la liste électorale tous les natifs de Nouvelle Calédonie ayant atteint l’âge de 18 ans, ainsi que tous les Calédoniens présents sur le territoire calédonien depuis au moins dix ans.

de nouveaux citoyens calédoniens à la liste électorale. On aurait pu prévoir cinq ans ou trois ans. On aurait pu aussi envisager que tout le monde vote. Le Gouvernement n’a pas fait ce choix et, sur ce point, la commission des lois lui a donné raison. Monsieur le ministre de l’intérieur, vous avez évoqué un amendement dont je suis l’auteur.

avec les parties calédoniennes, que la position que j’ai fait adopter par la commission des lois était jugée excessive et qu’on voulait en finir une fois pour toutes, non pas

à préférer l’accord à la recherche d’une solution unilatérale par le Parlement français. J’espère que ce compromis, que j’ai accepté, pourra prévaloir dans nos votes d’aujourd’hui. Au delà, un certain nombre d’autres questions se posent. En ce qui concerne le partage des sièges entre les provinces, le ministre de l’intérieur a dit que la revendication lui paraissait fondée, mais qu’il valait mieux la traiter dans le cadre d’un accord. Je partage son point de vue.

campagne le soir en mobilisant ses électeurs dans les meetings et négocier le matin pour trouver un accord avec ses adversaires. Si nous voulons vraiment un accord qui assure le temps long et la stabilité de la Nouvelle Calédonie, les élections doivent avoir lieu le plus tôt possible.

mes chers collègues, : respect et humilité. Nous sommes au rendez vous avec l’histoire, un rendez vous manqué… Le temps est venu de parler, de parler de ce qui constitue le cœur du pari de l’intelligence sur le devenir de mon pays, la Kanaky. Ce pari est le suivant : faire peuple. « Moi je suis passager, mais je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce que je peux faire pour que le pays que je lègue à mes fils soit le plus beau pays. » Voilà les mots de Jean Marie Tjibaou. Aujourd’hui, je veux pouvoir dire les miens, ceux d’une lutte, d’un espoir, d’un rêve qui anime ma chair, celle de mes aïeux, et maintenant celle de mes enfants et petits enfants. Ce rêve qu’on porte en nous et qui a été embrassé par les gens de ce pays : le rêve de la liberté de penser, dire et de faire en notre nom propre ! Nainville les Roches en 1983 en est le symbole. Je dis « symbole », car cette main tendue pèche à être prise. Je veux croire qu’elle le sera un jour par l’ensemble des communautés qui feront peuple en Kanaky.

Je veux exprimer la voix d’un peuple debout, qui existe, qui vit et qui crie haut et fort son existence, sa résistance. Le pari de l’intelligence était de construire une communauté de destin, autour du peuple kanak, avec les descendants de la colonisation dans un pays commun. Qu’en est il aujourd’hui de ce pari ? Ce projet de loi confirme l’adage « diviser pour mieux régner ». C’est une démarche meurtrière. La représentation nationale et le Gouvernement peuvent ils décider sans le peuple concerné ?

Dois je comprendre que nous sommes des menteurs ? Ou ce document existe t il réellement ? Je note tout simplement que la saisine du congrès de la Nouvelle Calédonie sur cette réforme constitutionnelle n’a pas été faite. Nous sommes déjà le 27 mars au pays ; ici on est le 26. Comprenez ceci : les décisions depuis Paris seront toujours en retard face à notre histoire, car le destin de notre peuple se dessine sur sa terre. Ce projet de loi s’inscrit à contresens de notre histoire. On vient toucher au cœur même de ce qui constitue la citoyenneté calédonienne : le corps électoral. Nous ne pouvons pas examiner ce projet de loi unilatéral sous l’unique prisme des valeurs républicaines si fondamentales pour la Nation française que sont l’universalisme et la démocratie.

depuis 1789 », laissant ainsi entendre que toute position contraire serait antidémocratique. À quelle forme de démocratie fait on référence ? Dois je vous rappeler, monsieur le ministre, moi qui suis Kanak,

1945 le gouverneur Jacques Tallec fut à l’origine du premier gel du corps électoral calédonien empêchant l’inscription des Kanaks ? Qu’en 1946, le ministre de la France d’outre mer de l’époque a proposé un projet de création d’un double collège électoral afin de séparer les électeurs kanaks des colons électeurs qu’il aura fallu attendre 1957 pour que l’Assemblée territoriale puisse véritablement représenter l’ensemble de la population non kanak et kanak ? Monsieur le garde des sceaux, dois je vous induite par la circulaire Messmer de 1972, qui a volé au peuple kanak sa légitimité et sa majorité démocratique ? Cela fait beaucoup de rappels historiques, mais ne dit on pas que la pédagogie est affaire de répétition ? Pour autant, nous éviterions bien volontiers une répétition des conséquences du passé. Au nom de la démocratie, le Gouvernement oublie son passé et brandit les valeurs républicaines à géométrie variable. On notera qu’en 2023, la Cour de cassation a considéré que tant que le pays était sur la voie de la décolonisation, il n’y avait pas de nécessité démocratique à faire évoluer le corps électoral. La réouverture du corps électoral ne fait que reprendre la stratégie de colonie de peuplement pour s’emparer une nouvelle fois du pouvoir. Le gouvernement français est il en mesure de considérer que la démocratie prime sur la décolonisation ? On a tout connu, tout subi, des soulèvements, des morts, mais le combat d’un peuple n’a pas de prix. Ce projet de loi est un héritage de la pensée coloniale, un héritage des méthodes d’antan qui ont réduit nos anciens au code de l’indigénat, les privant du droit de vote sur leur propre terre. Le consensus, par un accord global, est le seul et unique moyen de respecter notre histoire. Le gouvernement actuel passe en force sur ce qui est essentiel à la survie d’une communauté de destin. Le point 5 de l’accord de Nouméa indique tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette “irréversibilité” étant constitutionnellement garantie ». Or, aujourd’hui, aucun accord n’a été trouvé et le Gouvernement passe en force. Ce mode de fonctionnement dédaigneux, paternaliste et déconnecté de nos pays met en lumière le caractère profondément colonialiste de l’intervention de l’État dans le dossier calédonien. La conclusion d’un accord global est le chemin consensuel le plus approprié. On ne discute pas sous la menace. Le corps électoral est le ciment de la citoyenneté calédonienne. Rompre les équilibres trouvés, c’est volontairement éradiquer la notion de peuple kanak Cette réforme prévoit d’élargir le corps électoral à tous les résidents de plus de dix ans. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la circulaire Messmer, nous rendant minoritaires sur nos terres et laissant la maîtrise de nos administrations locales entre les mains des populations accueillies. C’est ainsi que le gouvernement français veut consacrer dans la Constitution la colonie de peuplement et légitimer la « minorisation » du peuple kanak : c’est légitimer pour mieux recoloniser. Par ailleurs, le gouvernement français rompt avec ses engagements internationaux. La Kanaky est inscrite depuis 1986 sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Le projet de loi est en contradiction avec le point 11 de la résolution de l’Assemblée générale des Les puissances administrantes devraient veiller à ce que l’exercice du droit à l’autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique dues à l’immigration ou au déplacement de populations dans les territoires qu’elles administrent. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir », disait Frantz Fanon. La nôtre est intergénérationnelle et nous voulons la remplir : celle de la lutte pour pour la pleine souveraineté. Nous sommes ici pour porter ce flambeau et personne ne nous l’enlèvera ; nos enfants le porteront à leur tour. Tant qu’il y aura un Kanak sur cette terre, la revendication subsistera. Aimé Césaire disait : « Faire un pas avec le peuple, pas deux pas sans lui.

La perte de la légitimité historique du peuple kanak nous fait revenir au temps que l’historien Louis José Barbançon dénommait « le pays sans nous ». D’un peuple kanak minoritaire à un peuple français majoritaire, il n’y a qu’un pas. Face à l’oppression, au mépris et à l’humiliation, mon peuple vous répond : respect et humilité. Le peuple français n’est pas l’ennemi du peuple kanak. Je ne suis pas venu dire que votre universalisme et votre démocratie sont meilleurs que notre droit d’exister. Chacun ses valeurs, chacun ses responsabilités. Je suis venu exprimer, sans haine ni mépris, notre droit de faire pays, tout comme vous aspirez à votre souveraineté. Pourquoi serions nous moins légitimes à parler de nous mêmes ? Le FLNKS, réuni en congrès ce samedi 23 mars, a réaffirmé son unité. À l’instar de l’ensemble des groupes progressistes et du groupe CRCE Kanaky, il demande le retrait de ce texte. Mesdames, messieurs les parlementaires, rejeter ce texte, c’est respecter le chemin de l’histoire. La

M. Xowie et ses collègues du groupe CRCE Kanaky proposent, par leur motion tendant à opposer la question préalable, que le Sénat n’examine pas le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle Calédonie. Nos collègues estiment, notamment, que le renoncement à ce texte ne serait pas de nature à créer un vide juridique pendant le temps que nécessitera la poursuite des négociations sur place. d’abord, relevons que le texte que nous présente aujourd’hui le Gouvernement ne prétend ni régler l’intégralité de la question de l’avenir institutionnel et politique du territoire ni même apporter le commencement d’une réponse globale.

Nous regrettons que cet objectif n’ait pas pu être atteint à ce stade, mais nous demeurons confiants en la possibilité d’aboutir à une feuille de route consensuelle vers un destin commun pour l’ensemble des citoyens de la Nouvelle Calédonie.

En l’occurrence, ce que le projet de loi constitutionnelle vise à faire, c’est pallier l’une des principales difficultés soulevées par l’arrivée à son terme théorique de l’armature juridique actuelle : la problématique des modalités d’inscription sur la liste électorale « spéciale

Plus encore, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, le constituant a fait prévaloir l’interprétation d’un corps électoral « gelé » à l’article 77 de la Constitution.

qu’aux articles 1 et 3 de la Constitution et, enfin, à l’article 3 du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont admis la validité de limitation du corps électoral au regard de ces différents principes, c’était strictement à condition que cela s’inscrive dans un cadre temporel transitoire et donc limité dans le temps. Ce cadre découle du processus défini par l’accord de Nouméa, auquel la Constitution fait par ailleurs explicitement référence, et a prévu par conséquent un titre spécifique pour la Nouvelle Calédonie dont les dispositions sont transitoires. Après l’organisation des trois consultations d’autodétermination, et comme l’a fait valoir le Conseil d’État, nous sommes arrivés au terme du processus, sa mise en œuvre devant être regardée comme étant désormais complète. Il nous appartient donc de tirer toutes les conséquences de l’achèvement de ce processus. Le rapporteur de l’Assemblée nationale l’avait par ailleurs fait valoir dès l’examen du texte constitutionnel relatif à la Nouvelle Calédonie de 2007, en rappelant qu’« après le référendum d’autodétermination, quel qu’en soit le résultat, un nouveau régime devra être défini pour le corps électoral Je ne voudrais pas terminer cette intervention sans rappeler que le risque juridique n’est pas mince. Il ne serait pas responsable d’organiser des élections sans avoir la garantie de la régularité de leurs fondements juridiques. Cette se double d’une réalité changeante sur le terrain, accroissant d’autant plus son acuité. L’évolution de la démographie de la Nouvelle Calédonie depuis les années 1990

Désormais, plus de 42 000 électeurs sont ainsi écartés du vote pour la gouvernance du territoire calédonien. Enfin, ce projet de loi s’inscrit dans une démarche subsidiaire à tout accord futur il ne traite que d’une seule question, qui demande une réponse juridique rapide, faute de quoi la démocratie calédonienne se retrouverait suspendue, ce que personne ne souhaite. Ce texte ne préempte pas les négociations autour de cet accord ; il nous permet de nous prémunir d’une absence d’accord sur un point unique, celui de l’organisation régulière des prochaines élections provinciales. L’ensemble des autres sujets intéressant l’avenir de la Nouvelle Calédonie, tout comme ce corps électoral, pourront toujours faire l’objet d’un accord qui fera alors évoluer le droit applicable. Le législateur national y sera prêt. Permettre à un tel accord d’interrompre l’entrée en vigueur du texte s’il venait à être voté par le constituant est l’objet même du mécanisme proposé par le Gouvernement à l’article 2, même si, nous le verrons, une souplesse supplémentaire doit lui être apportée.

possible en Nouvelle Calédonie sans que les Calédoniens s’entendent eux mêmes sur leurs institutions, leur avenir et la manière dont s’exercera dans le futur le droit à l’autodétermination. En effet, celui ci ne disparaît pas

province et au congrès de Nouvelle Calédonie puissent se tenir et qu’elles ne soient pas retardées. C’est en effet seulement après ces élections que le maximum de chances réapparaîtra pour la conclusion d’un accord.

demande que des travaux soient menés en concertation avec les services de l’État afin d’évaluer les impacts et réaliser des projections sur l’évolution de ce corps électoral en prévision des élections provinciales de 2024. » Et ledit document est signé, je

un ensemble d’îles au climat presque idéal, bordées de plages avec des palmiers, au milieu d’une eau d’un bleu sans pareil, au sein d’un lagon parmi les plus grands du monde, protégé par une incroyable barrière de corail…

l’envers de ce décor. Sur ce même archipel, qui compte environ 270 000 habitants, 42 000 personnes sont privées du droit de vote, soit près de 20 % de la population. Imaginez donc vivre là bas depuis vingt cinq ans, travailler, payer vos impôts, ou même y être né, et être privé du droit démocratique le plus basique et fondamental, privé de votre statut de citoyen, privé du droit de choisir ceux qui vous gouvernent et qui décident de l’avenir de votre territoire

En 1998, le corps électoral a d’abord été restreint par l’accord de Nouméa aux personnes inscrites sur les listes électorales jusqu’en 1998 et aux personnes arrivées après 1998

C’est ainsi que seules peuvent voter aux élections territoriales les personnes inscrites sur les listes jusqu’en 1998. Cette situation, inimaginable pour un Français de l’Hexagone, a été acceptée à l’époque en raison de son caractère transitoire. ans plus tard, l’accord de Nouméa est caduc : à trois reprises, lors des référendums de 2018, 2020 et 2021, la population calédonienne a exprimé sa volonté de rester française.

celui ci serait restreint aux personnes inscrites sur la liste électorale générale de Nouvelle Calédonie, qui y sont nées ou domiciliées depuis au moins dix ans. L’adoption de ce texte permettra à 25 000 personnes supplémentaires de participer aux prochaines élections provinciales. C’est un juste rééquilibrage.

Il faut dire la vérité : même si nous y sommes tous favorables, la perspective de parvenir à un accord avant les élections est très incertaine. Le dégel du corps électoral est une première étape pour un retour vers un processus démocratique acceptable. il doit être assorti d’un rééquilibrage de la représentativité des trois provinces. En effet, la situation économique et un fort tropisme vers la province Sud ont modifié la répartition de la population sur le territoire.

Sans cela, nous enverrions un très mauvais message aux autres territoires ultramarins, et même à certains territoires de l’Hexagone. Par trois fois, la Nouvelle Calédonie a réaffirmé son choix d’être française. Il est donc de notre responsabilité de rétablir un véritable processus démocratique sans lequel les discussions futures seraient impossibles.

que notre rapporteur Philippe Bas propose de procéder à un dégel uniquement pour les élections de 2024. Nous examinerons donc le sous amendement du président de la commission des lois visant à revenir sur cette modalité.

que les dispositions ayant suscité l’accord de tous les partenaires au travers des accords de Nouméa et de Matignon. Il nous paraissait donc quelque peu gênant de constitutionnaliser des dispositions n’ayant pas fait l’objet d’un accord général.

un aspect majeur de la définition de sa citoyenneté, un questionnement profond sur la légitimité politique et historique de la décision que nous nous apprêtons à prendre

Opposer les principes démocratiques républicains à ceux qui commandent au respect du droit à l’autodétermination des peuples colonisés est par nature inconséquent et intenable. Personne ne le conteste, pas même les indépendantistes. Les restrictions du corps électoral excluent d’année en année davantage de citoyens et de citoyennes. Le corps électoral doit être réformé : tout le monde le reconnaît. Peut être toutes les parties concernées pourraient elles tolérer l’unilatéralité, si la réforme était parfaitement consensuelle et d’ordre purement technique ; mais c’est tout le contraire. Cette réforme touche au cœur sensible du sujet. La question du corps électoral est intimement liée au fait que la Nouvelle Calédonie a été une colonie de peuplement. En 1972, Pierre Messmer, alors Premier ministre, écrivait : « La revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. » Pour cela, il proposait « l’immigration massive de citoyens français métropolitains ». ». C’est pourquoi la question du corps électoral a toujours été au cœur de toutes les discussions. C’est pourquoi elle est consubstantielle à la question de la citoyenneté calédonienne. C’est pourquoi, aussi, en 2017, nous avons gelé par un accord constitutionnel, comme une promesse de l’État de son engagement sans faille à respecter le contrat social issu de l’accord de Nouméa. Or, depuis 2020, nous avons multiplié les fautes.

du fait de l’épidémie. Ensuite, lorsque Sonia Backès, cheffe de file des loyalistes, a été nommée secrétaire d’État. Quelle idée ! Comment dire plus clairement que ce gouvernement n’entend plus être impartial ? Aujourd’hui, enfin, lorsqu’il nous est demandé de prendre le risque de trop remettre en cause la parole de l’État en rompant, unilatéralement, le contrat de 1998, et « détricoter les principes qui […] avaient assuré la paix civile », comme le décrit Jean François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard pour les outre mer, dans une tribune publiée dans.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question du corps électoral est politiquement cruciale en Kanaky comme en Nouvelle Calédonie.

Le motif invoqué est que le corps électoral citoyen du pays « ne répond plus aux exigences démocratiques résultant de nos principes constitutionnels et des engagements internationaux de la France » : « Au regard de cette réforme et des délais nécessaires à sa mise en œuvre, il apparaît ainsi nécessaire de repousser le renouvellement de repousser le renouvellement des assemblées. » Le Gouvernement veut ainsi ouvrir le périmètre du peuple calédonien aux arrivants français résidant depuis dix ans sur le territoire. Ce corps électoral, devenu glissant, organise de fait la noyade démographique du peuple kanak. C’est le grand remplacement… Par ailleurs, ce corps électoral glissant est contraire aux résolutions de l’ONU et met fin aux équilibres patiemment négociés en 1998. De fait, il alimente pour certains l’idée de rupture frontale avec le principe même du processus de décolonisation. Le projet, uniquement justifié par la révision constitutionnelle unilatérale, est la négation même des accords de Matignon et de Nouméa. L’État partial tire un trait sur le processus de décolonisation en Nouvelle Calédonie. Il met à mal plus de trente ans d’efforts pour parvenir à construire une citoyenneté calédonienne légitime aux yeux de tous, fruit d’un compromis historique entre des partenaires calédoniens fidèles aux idéaux de réconciliation symbolisés par la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean Marie Tjibaou. Le passage en force du Gouvernement sous la forme d’une réforme à marche forcée, avec notamment un ultimatum au 1 juillet, est en totale contradiction avec la méthode privilégiée par les précédents gouvernements, qui ont choisi le dialogue et le consensus auprès des partenaires locaux pour parvenir à deux accords de paix. Tout le monde ici se souviendra que les accords de Matignon et de Nouméa auront permis de déployer le vivre ensemble pendant trente six années paisibles. Le Gouvernement prend donc une très lourde responsabilité en engageant cette réforme unilatérale, avec la caution des parlementaires que nous sommes si le texte venait à être adopté en l’état. Pourquoi un tel empressement, pourquoi un passage en force, alors que rien ne le justifie ? Il y a, comme chacun sait, des discussions en cours entre les partenaires calédoniens. D’ailleurs, les indépendantistes doivent discuter parallèlement avec deux tendances loyalistes qui refusent de négocier ensemble. Les indépendantistes Les indépendantistes affirment qu’ils n’ont jamais été opposés à l’arrivée de populations nouvelles, nécessaires pour asseoir un développement économique ambitieux. Néanmoins, ils souhaitent préserver le corps électoral tant que le processus d’émancipation n’a pas abouti. Rappelons d’ailleurs que dès 1983, à Nainville les Roches, les indépendantistes avaient ouvert la citoyenneté calédonienne aux autres communautés arrivées par la colonisation. Aujourd’hui, ils ne sont pas opposés à l’intégration des natifs, actant ainsi le principe du droit du sol, mais ils considèrent que toutes ces questions doivent être traitées dans le cadre d’un accord global. Seule cette solution saura garantir une paix civile durable ainsi qu’une stabilité politique, économique et sociale.

Seule la conclusion d’un accord global peut assurer et garantir la continuité des deux accords de paix conclus entre partenaires calédoniens. Je salue

la continuité du vivre ensemble. Il offre, s’il en était besoin, une perspective salvatrice : celle du respect de la parole donnée de la République à l’ensemble

Aujourd’hui, nous avons l’occasion d’écrire un nouveau chapitre institutionnel et politique, à condition de ne pas renier l’esprit de consensus trouvé voilà maintenant plusieurs décennies. Ces accords ont ouvert la possibilité de ne faire voter, pour certaines élections, que ceux qui pouvaient justifier d’une résidence continue pendant au moins dix ans avant 1998. termes, ces accords ont restreint l’accès au suffrage d’une partie des Calédoniens pour préserver la paix. Une restriction unique du droit français, constitutionnalisée par les « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle

Cette situation permettra à 25 000 Calédoniens de participer aux prochains scrutins locaux dès le mois de décembre prochain. Comme l’a rappelé le rapporteur, après la période du 1 juillet 2024, les citoyens installés continuellement sur l’archipel depuis 2014 pourront voter aux prochaines élections locales.

Nous le savons, l’inscription d’une partie des citoyens sur une liste spéciale revient à reconnaître l’existence d’une citoyenneté néo calédonienne. Au moment des accords de Nouméa, ce principe représentait la pierre angulaire des accords entre loyalistes et indépendantistes. Il s’agissait de reconnaître la spécificité de ce territoire, son histoire et la représentativité de son peuple premier. C’est d’ailleurs une exigence des Nations unies. D’un côté, les indépendantistes accueillaient les Européens avec un « statut de résident ». De l’autre, les loyalistes acceptaient que seuls les résidents installés depuis bien plus longtemps accèdent à certains scrutins. Aussi ne faudrait il pas que ce dégel apparaisse, aux yeux des indépendantistes, comme une victoire des loyalistes. Une telle situation pourrait replonger l’archipel dans un long cycle de violence. Outre ces considérations politiques, il ne faut pas s’habituer à ce que de telles entorses démocratiques perdurent.

Au delà du contexte, nous sommes attachés à ce qu’un dialogue impartial, loyal et intransigeant demeure entre toutes les parties. Par ailleurs, l’avenir de l’archipel ne doit pas se faire sans la mise en place d’une coopération renforcée avec le Caillou dans les secteurs économique, énergétique et social. Il ne doit pas non plus s’opérer au détriment de la stabilité régionale. L’autodétermination est une très grande inconnue dans l’équation géopolitique de l’Indo Pacifique, dont je rappelle que le plus gros problème est la politique impérialiste du gouvernement chinois. Pour toutes ces raisons, nous attendons beaucoup du débat qui s’offre à nous. Pour le moment, ce que nous souhaitons par dessus tout, je le répète, c’est l’assurance de garanties permettant de préserver l’archipel d’une nouvelle crise. La parole

À cet égard, signalons que le nouveau report de la signature du pacte sur le nickel n’est évidemment pas un bon signal. Défi social, ensuite, avec des inégalités encore plus marquées qu’en métropole. Ainsi, plus de 50 000 habitants sur 270 000 vivent sous le seuil de pauvreté et la population est confrontée à la cherté des prix.

Défi politique, enfin, avec la nécessité de définir, après presque quarante ans de paix civile, les voies et moyens permettant d’aboutir à la définition d’un destin commun, partagé par tous les Calédoniens. Le retard pris dans la définition de ce destin commun touche directement les autres sujets – économique, social, financier –, d’autant qu’il prolonge une période d’incertitude inhérente à la tenue des trois consultations prévues par l’accord de Nouméa. Bien évidemment, la vie démocratique doit se poursuivre pendant cette transition et les élections provinciales doivent se tenir dans les meilleures conditions possible. C’est le sens du report de quelques mois de la consultation électorale provinciale, Il s’agit aujourd’hui de permettre que ces élections se tiennent régulièrement par le dégel du corps électoral. Cela suppose d’intégrer dans le corps électoral élisant les conseillers des provinces des citoyens nés ou arrivés en Nouvelle Calédonie après 1998.

loi constitutionnelle est absolument indispensable au regard du principe de l’égalité du suffrage. Bloquer encore l’évolution du corps électoral poserait non seulement un problème démocratique, mais aussi, et surtout, une difficulté juridique. En effet, les élections se font bien évidemment sous le contrôle du juge. Le Conseil d’État a d’ailleurs envoyé un message très clair en indiquant qu’une consultation électorale qui se tiendrait sur la base d’une liste électorale arrêtée en 1998 serait frappée d’irrégularité, en raison non seulement d’engagements internationaux, mais aussi de la Constitution. Le dégel du corps électoral est donc aujourd’hui non pas une option politique, mais une nécessité juridique.

Puisqu’il nous faut bien avancer pour garantir la régularité juridique des prochaines élections provinciales, le Gouvernement nous propose de retenir une durée de résidence minimum de dix ans en Nouvelle Calédonie pour les nouveaux électeurs et, ainsi, un corps électoral glissant, et non plus gelé. Cette Cette proposition nous paraît raisonnable en ce qu’elle permet de s’assurer d’un lien suffisamment fort et constant entre le nouvel électeur et la Nouvelle Calédonie. Elle ne remet donc en cause ni l’existence d’une spécificité propre au territoire calédonien en matière électorale, avec l’existence d’un corps restreint, ni même le principe d’une citoyenneté calédonienne. Cette proposition ne semble pas susciter d’opposition marquée du côté des loyalistes comme du côté des indépendantistes. elle n’est pas de nature à compromettre la conclusion d’un accord global sur l’avenir politique et institutionnel. Cependant, afin de ne pas préempter les conclusions de cet accord qui doit intervenir entre les parties calédoniennes, l’État doit selon nous intervenir le moins possible de manière unilatérale. Nous avons ainsi bien conscience que l’adoption de ce texte constitue une exception dans le mode d’action de l’État, que seules l’urgence et la contrainte juridique impérieuse liée à la régularité des élections à venir viennent justifier et sous la réserve qu’un accord n’ait pas été conclu avant le 1 juillet prochain. L’État doit en effet demeurer

monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis l’accord de Nouméa en 1998 que l’on doit à Lionel Jospin, seuls peuvent voter aux élections provinciales et du congrès les personnes et leurs descendants qui remplissaient les conditions pour voter au référendum approuvant cet accord. a t elle été décidée à l’époque ? L’accord de Nouméa prévoyait la reconnaissance d’une citoyenneté calédonienne au sein de la citoyenneté française. Cela correspondait au point d’équilibre des aspirations des Néo Calédoniens sur leur personnalité : l’identité kanake, la citoyenneté calédonienne, la nationalité française. Cette citoyenneté comporte deux traductions dans l’accord de Nouméa : les limitations apportées au corps électoral et les mesures pour préserver l’emploi local. C’est en 2007 que ce corps électoral restreint a été gelé par une révision constitutionnelle décidée par le Président de la République Jacques Chirac. Le corps électoral restreint était un engagement pris dès les accords de Matignon ; nous pouvons d’ailleurs dire aujourd’hui que c’était la condition d’une décolonisation réussie. Aujourd’hui, le gel du corps électoral exclut du suffrage des natifs de Nouvelle Calédonie, y compris des Kanaks, mais aussi des personnes installées depuis de nombreuses années. Aussi, il nous paraît légitime de modifier la composition du corps électoral, mais pas n’importe comment. En 1984, un statut de la Nouvelle Calédonie est adopté sans tenir compte des revendications des indépendantistes sur le corps électoral. Ce sera l’un des éléments déclencheurs du boycott actif des élections territoriales de novembre 1984, puis des « événements » qui lui succèdent.

Aujourd’hui, quarante après, on retrouve conjugués les deux éléments déclencheurs de 1984 et 1988 : le corps électoral et le calendrier. Cette situation est aggravée par un autre facteur, la volonté du Gouvernement de passer en force, qui met une pression insupportable sur les représentants politiques locaux.

constitutionnelle comprend deux mesures que l’on pourrait qualifier de baroques. Non seulement il fait de la révision constitutionnelle une réforme par défaut, mais surtout il méconnaît les droits du Parlement en déléguant au pouvoir réglementaire les modalités d’application de la révision.

Cet ultimatum n’est pas acceptable. Le Gouvernement enchaîne les fautes depuis le départ du Premier ministre Édouard Philippe : organisation à marche forcée du troisième référendum, remise en cause de l’impartialité de l’État avec la nomination de Sonia Backès, modification unilatérale du corps électoral ce projet de loi constitutionnelle, nomination de rapporteurs partiaux à l’Assemblée nationale, remise en cause de la parole de l’État donnée lors de l’accord de Nouméa. C’est une pente dangereuse que vous prenez là, monsieur le ministre. Le rôle de l’État français doit être celui d’un partenaire actif, mais toujours impartial ; il doit faciliter l’émergence d’un accord global sur une nouvelle organisation politique et institutionnelle. Modifier le corps électoral, oui. C’est une nécessité constitutionnelle. Pour autant, ce n’est pas aujourd’hui une urgence institutionnelle. En profiter pour modifier la répartition des sièges au congrès et aux assemblées des provinces, non. Cette répartition, qui remonte aux accords de Matignon, est un pilier du compromis historique qui a ramené la paix civile. Toute modification n’est envisageable que dans le cadre d’un futur accord politique global. Vous le savez, la situation locale est difficile : le territoire connaît une crise économique et sociale, la filière du nickel est en grande difficulté, l’usine du Nord est à l’arrêt, les effets économiques en cascade paralysent presque tous les secteurs d’activité, les déficits sociaux s’aggravent.

au service de la poursuite d’une décolonisation réussie. Il est encore temps de prolonger la poignée de main entre Tjibaou et Lafleur et de parvenir à un destin commun.

à des milliers de Calédoniens de participer à la vie démocratique de la Nouvelle Calédonie. Quelle est la situation aujourd’hui ? Plus de 20 % des 220 000 électeurs en Nouvelle Calédonie sont privés du droit de vote aux élections provinciales.

Parce qu’ils sont arrivés en Nouvelle Calédonie après le mois de novembre 1998 ou parce qu’ils sont nés de parents installés après cette date couperet, des milliers de Calédoniens, de cœur ou de naissance, qui y ont passé toute leur jeunesse et qui y construisent leur avenir, sont exclus de la vie démocratique de notre territoire. Mes chers collègues, jamais ni les accords de Matignon ni l’accord de Nouméa n’ont fixé les conditions d’un tel gel du corps électoral. Aucun texte soumis à l’approbation des Calédoniens n’a gravé dans le marbre cette date couperet de novembre 1998. ce gel a été ajouté postérieurement, par la révision constitutionnelle de février 2007. De plus, cette disposition n’a été intégrée que dans la perspective des élections provinciales de 2009 et de 2014, pour permettre aux scrutins d’autodétermination de se dérouler dans le calme. Il s’agissait donc d’une disposition transitoire, qui, hélas ! perdure déjà depuis trop longtemps. Dégeler le corps électoral de la Nouvelle Calédonie pour permettre un retour de la démocratie est donc une nécessité absolue. Au delà de cet aspect démocratique, ne pas dégeler le corps électoral reviendrait à nous placer en dehors des exigences constitutionnelles et conventionnelles qui nous lient, ce qui ne serait tenable ni juridiquement ni politiquement. Enfin, mes chers collègues, ne pas voter ce texte reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. Comment imaginer que les élections provinciales qui se tiendront au mois de décembre prochain ne soient pas contestées par les Calédoniens ? Comment imaginer que les nouvelles assemblées des provinces et du congrès soient pleinement légitimes si 20 % des électeurs sont tenus à l’écart des urnes ? Nous ne pouvons le concevoir. En ce sens, le groupe Les Républicains votera avec vigueur en faveur de l’article 1 permettant de dégeler le corps électoral des élections provinciales pour toute personne née en Nouvelle Calédonie ou y résidant depuis au moins dix ans. Cela permettra à près de 25 000 Calédoniens, aujourd’hui exclus, de s’exprimer dans les urnes à l’occasion du prochain renouvellement des assemblées de province et du congrès. Je serai particulièrement vigilant à ce que ce dégel soit ferme et définitif.

de réduire de moitié, soit à cinq ans, la durée de résidence nécessaire pour faire partie de cette liste électorale. Nombreux sont les Calédoniens qui épousent un métropolitain ou un Ultramarin du Pacifique ou d’ailleurs avec le souhait de fonder une famille. Il me semble qu’une telle disposition serait une mesure de justice et une marque de confiance à l’égard de ceux qui ont adopté la Nouvelle Calédonie comme territoire de cœur. En retour, celle ci se doit de les accueillir et de les intégrer. Le second amendement a un objet au moins aussi fondamental que le dégel du corps électoral prévu par ce projet de loi constitutionnelle dans sa version initiale. Il vise à rétablir le principe de l’égalité devant le suffrage en Nouvelle Calédonie en rééquilibrant la répartition des sièges des provinces au sein du congrès. Les accords de Matignon, il y a trente six ans de cela, puis l’accord de Nouméa, dont je rappelle qu’il était transitoire, ont fixé la répartition des sièges au congrès de la Nouvelle Calédonie. Cette répartition donnait déjà un avantage de représentativité aux provinces à majorité indépendantiste : Nord et îles

Cette exception démocratique donne ainsi aux habitants de la province des îles Loyauté une représentativité plus de deux fois supérieure à celle des habitants de la province Sud. Au regard du principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, de tels écarts ne sont plus acceptables. Rééquilibrer la répartition des sièges au congrès est donc indispensable pour que cette révision constitutionnelle permette véritablement de remettre la démocratie au cœur du fonctionnement institutionnel de la Nouvelle Calédonie. À ceux qui, aujourd’hui, seraient tentés de s’abstenir et de préférer l’excès de prudence, je dis : ne cédez pas au chantage à la paix, qui, en plus d’être démocratiquement dangereux, ne fait pas honneur au destin commun que tous les Calédoniens s’efforcent de bâtir depuis trois décennies. Ce n’est pas l’excès de prudence, mais bien les actes et la volonté qui donneront à la Nouvelle Calédonie la force de relever les défis qui l’attendent. Mes chers collègues, c’est de l’avenir de la Nouvelle Calédonie qu’il est question et c’est de cet avenir que je désire vous parler. Depuis ce 26 juin 1988 où Jean Marie Tjibaou et Jacques Lafleur se sont serré la main à Matignon, afin que tous les Calédoniens puissent avancer ensemble vers un destin commun, la Nouvelle Calédonie a fait la preuve de sa volonté et de sa détermination à concevoir l’avenir. Un avenir où chaque Calédonien trouvera sa place au sein de la société. Un avenir où chaque culture pourra s’exprimer dans sa beauté, sa richesse et sa diversité. Un avenir où, ensemble, nous relèverons les défis économiques qui se dressent devant nous. Un avenir commun pour la Calédonie et pour les Calédoniens au sein de la République française, ainsi qu’ils l’ont décidé majoritairement à trois reprises. collègues, avec force, je vous demande de voter en faveur de ce projet de loi constitutionnelle et de soutenir les amendements que je présenterai. Il y va de l’avenir de la démocratie calédonienne, de son avenir dans la République et de ce destin commun qui, plus que jamais, nous est si cher.

monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui, sur fond de crise économique et sociale, du dégel du corps électoral en Nouvelle Calédonie. Les négociations sur cet enjeu constituent l’une des pierres angulaires de l’édifice de la paix. Rappelons que, au moment des accords de Matignon, la Nouvelle Calédonie était au bord de la guerre civile. Michel Rocard, en tant que Premier ministre, devait relever des défis majeurs : ramener la paix, retisser les liens de la confiance et engager un mouvement de décolonisation pacifique et viable. Les accords de Matignon ont assuré pendant dix ans le maintien d’une paix civile et engagé la réconciliation. La Nouvelle Calédonie s’est organisée autour de trois provinces, pour donner aux Kanaks la responsabilité politique des régions où vivent la majorité d’entre eux et favoriser leur développement économique. Le rééquilibrage entre les communautés et les territoires a progressé, appuyé par un effort financier sans précédent de l’État au profit des équipements publics et par un programme de formation. La culture kanake est désormais reconnue. Le magnifique centre culturel Tjibaou, l’un des grands travaux du président Mitterrand, en est un témoignage patent. À mon tour, je tiens à saluer, dans le même élan, le courage politique de Jacques Lafleur. L’accord de Nouméa, œuvre de Lionel Jospin en 1998, a poursuivi ce mouvement. Il exprime une vision partagée de l’histoire et de l’avenir du pays. Pour la première fois, l’État et les partis politiques de la Nouvelle Calédonie portent un regard commun sur la période douloureuse, très douloureuse, de la colonisation.

La paix, c’est la négociation, c’est le courage de céder sur certains points au nom d’un objectif plus essentiel, le courage de transformer l’ennemi en interlocuteur. La méthode éprouvée par Michel Rocard, puis par Lionel Jospin, doit nous inspirer. Elle a affirmé la volonté de l’État de trouver par la négociation une solution de compromis, dans laquelle personne ne renierait ses idéaux.

Notre devoir est d’entretenir le travail accompli. En effet, la construction originale qui a été imaginée avait pour but de bâtir un destin commun pour la population pluriethnique néo calédonienne, constituée du peuple d’origine et de ceux qui, depuis cent soixante dix ans, s’y sont installés durablement. Le débat que nous avons aujourd’hui ne concerne pas seulement les Néo Calédoniens. Le débat qui nous amène est celui de la décolonisation, de l’autodétermination et du droit à l’émancipation. En érigeant l’accélération en système, l’exécutif se trompe. Cette marche forcée, dont nous faisons régulièrement les frais, le mène à une forme de brutalité institutionnelle. Les réformes rejetées par l’ensemble des citoyens se font désormais à coup de 49.3. Pour la Pour la situation de la Nouvelle Calédonie, la verticalité n’a pas sa place. Pourtant, alors que tous les acteurs en présence préconisent un accord global – même ici, au Sénat, et c’est heureux – et non partiel, vous avez fait le choix de scinder les sujets.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, c’est bien une nouvelle page qu’il nous revient collectivement d’écrire aujourd’hui, après que, à trois occasions, de trois référendums, nos compatriotes de Nouvelle Calédonie ont réaffirmé leur attachement à la France, ainsi qu’à notre communauté de destin.

596 personnes sont exclues du corps électoral. Dès lors, il est difficile d’imaginer priver nos concitoyens de participer à la désignation de la gouvernance de leur territoire.

du statut de la Nouvelle Calédonie sur la base de cet accord, qui aurait nécessairement comporté un volet consacré à la question du corps électoral. Malheureusement, si nous sommes ici aujourd’hui, c’est bien pour constater qu’il n’y a pas eu

du corps électoral gelé vers un système plus souple et, surtout, plus respectueux des exigences démocratiques. Si la durée de la présence préalable requise peut être discutée

la conclusion rapide d’un accord entre les acteurs calédoniens, seule manière d’aboutir à un règlement durable et global des problématiques de la Nouvelle Calédonie.

d’impartialité pour la tenue du troisième référendum. Oui, c’est vrai, les indépendantistes ont demandé le 8 avril 2021 l’organisation d’un référendum sur l’indépendance. La covid est arrivée en Nouvelle Calédonie en septembre 2021 – c’est la date du premier

si elle le peut. Mais, monsieur le ministre, vous qui faites de la politique, vous êtes assez intelligent pour comprendre que, six mois après avoir refusé de reporter de quelques mois un référendum, nommer au Gouvernement une personne qui représente l’un des camps a été perçu comme

nous devons écouter tous les Néo Calédoniens et favoriser leur accord pour un destin commun dans un cadre démocratique, évidemment. La Constitution est malheureusement impuissante à garantir cette qualité personnelle chez tous ceux qui peuvent contribuer à l’avenir de la Nouvelle Calédonie. Ce n’est pas son rôle, d’ailleurs, et cette disposition purement incantatoire n’a pas sa place dans un texte constitutionnel. C’est pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, tout en approuvant l’exigence impérieuse de l’impartialité de tous. Quel est l’avis du Gouvernement ? Il est

de la Nouvelle Calédonie, caricaturer les propos des uns des autres ou faire des amalgames avec des formations politiques qui n’ont aucun rapport.

la discussion générale. En effet, nous pensons que la méthode suivie est mauvaise. Il ne s’agit pas de remettre en cause la nécessité de définir un corps électoral qui soit conforme à notre Constitution pour tenir des élections. Nous avions voté pour le projet de loi

si vous sortez des négociations la question essentielle du corps électoral, qui est consubstantielle à la définition de la citoyenneté calédonienne, vous mettez en danger la possibilité même d’obtenir un accord

unilatérale, qui s’appliquerait en l’absence d’accord. Nous considérons qu’il faut faire l’inverse : d’abord essayer d’obtenir un accord, puis le ratifier. Vous pensez, monsieur le ministre, qu’en procédant de la sorte vous facilitez

de l’ensemble des parties avec le gouvernement français sur le destin commun des Calédoniens. Et, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, cet accord est le seul gage de stabilité pour l’avenir de la Nouvelle Calédonie. Imaginons que les élections n’aient pas lieu

la loi organique puisse reconduire le système mis en place pour les élections de 2024. des réactions que nous avons enregistrées en Nouvelle Calédonie et d’un débat qui s’est développé au sein de la commission et à l’intérieur du groupe

Nous avons tous pu prendre connaissance de l’injonction adressée par le député Nicolas Metzdorf au président Bruno Retailleau à cet

est à M. Georges Naturel. Je dispose malheureusement de peu de temps pour exposer la situation si singulière à laquelle cet amendement tend à remédier.

Cette répartition sur une base essentiellement démographique accordait un avantage aux provinces du Nord et des îles Loyauté, à majorité indépendantiste. Toutefois, le temps a passé et l’écart de population s’est grandement creusé, de sorte que la province Sud ne dispose que de 60 % des élus pour 75 % de la population totale de Nouvelle Calédonie. Alors qu’un membre du congrès élu dans la province Sud représente plus de 6 300 habitants, un élu de la province des îles Loyauté n’en représente que 2 600.

Mes chers collègues, parce qu’elle est indispensable au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, je vous invite donc à soutenir massivement cette initiative.

un élu. En septembre 1985, lors de la mise en place des régions dans le cadre du statut Fabius Pisani, le Conseil constitutionnel avait censuré un rapport de représentativité de 2.

tout à fait

Il faut que les élections puissent avoir lieu, donc que la question du corps électoral soit traitée et que la révision constitutionnelle aboutisse. Tout à l’heure, lorsque nous avons eu à examiner le sous amendement présenté par M. Buffet,

son amendement, en retenant cette rédaction : « Par dérogation à l’article 77 de la Constitution, la répartition des sièges entre les provinces au sein du congrès de la Nouvelle Calédonie

monsieur le ministre, que nous ayons un désaccord ! Celui ci est fondamental. Je me permets de vous dire qu’il s’agit de la liste électorale et non pas du décret de convocation des électeurs. Ce sont deux choses différentes

conjointe des présidents des deux assemblées. Ces derniers ne sont pas partie prenante à l’accord ; ils sont indépendants, comme l’est le Conseil constitutionnel. Par conséquent, il nous paraît souhaitable que ce soit eux, plutôt que la juridiction, qui prennent cette décision de constatation.

Les amendements n 17 et 33 ont tous deux pour objet de reporter au 1 juillet 2025 l’entrée en vigueur de cette loi constitutionnelle. Cela rendrait impossible la tenue des élections

des deux propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’espace réservé de son groupe le jeudi 11 avril prochain. Nous examinerions ainsi d’abord la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole,